jouent un rôle structurel dans l'organisation territoriale de la santé. Les communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, les centres de santé et les maisons de santé sont ainsi profondément liés aux ARS des territoires sur lesquels ils sont implantés.

les contours proposés dans la rédaction actuelle de cet article sont beaucoup trop vagues pour être validés en l'état. L'habilitation à agir par ordonnance accordée au Gouvernement laisse craindre des prises de décisions déconnectées des territoires.

à l'ingénierie pour les projets qu'ils portent et, surtout, des cofinancements pérennes. Ils considèrent, par ailleurs, que la structuration actuelle des ARS les éloigne de l'échelon territorial de proximité que représentent les communes et les intercommunalités. Cet amendement vise donc à favoriser la mise en place d'un partenariat

Les communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, et les projets territoriaux de santé sont des moyens de consolidation de l'exercice coordonné. Il serait pertinent de garantir l'accès et la participation à ces structures de l'ensemble des acteurs de santé, les médecins généralistes libéraux et les associations de médecins généralistes libéraux qui exercent en cabinet ou en visite. Tel est l'objet du présent amendement, qui tend à s'inscrire dans une dynamique de décloisonnement à tous les niveaux, notamment entre secteurs public et privé, afin d'améliorer la qualité, la sécurité et la pertinence des soins dispensés.

Vous le savez, ce plan porte l'ambition de faire de l'exercice coordonné le cadre de référence pour l'ensemble des professionnels de santé de ville à l'horizon 2022. L'article 19 de ce projet de loi y contribue, en offrant aux professionnels le bon encadrement juridique pour ce travail en commun, quelle que soit sa forme : CPTS, maison de santé pluriprofessionnelle- MSP -, ou centre de santé. La commission des affaires sociales a supprimé une disposition de cet article prévoyant que le statut de société interprofessionnelle de soins ambulatoires, ou SISA, autorise l'emploi et la rémunération par les MSP de professionnels, parmi lesquels les assistants médicaux.

En particulier, en sus de l'emploi direct par le médecin concerné, le recrutement et le salariat par une maison de santé constitue l'une des modalités qu'il convient de permettre, sans pour autant l'imposer. Cette disposition sert les médecins

de revenir sur l'amendement adopté par la commission des affaires sociales ; à défaut, nous empêcherions les maisons de santé pluriprofessionnelles d'employer, sous leur statut de SISA, un assistant médical.

soucieuse de défendre les apports du Sénat à ce texte, elle ne souhaite pas leur suppression. S'agissant plus particulièrement des ARS, si l'on peut regretter la relative imprécision de la demande d'habilitation, je partage la préoccupation exprimée par la commission des affaires sociales, dès 2014,

les centres de santé ont déjà vu leur statut refondu par ordonnance en 2018. Toutefois, il est cohérent de les inclure dans cette habilitation, qui concerne l'ensemble des formes d'exercice coordonné, dont ils font pleinement partie. Il s'agit, par exemple, de rendre possible

tend à modifier le sens de l'habilitation à prendre par ordonnance des mesures pour définir des structures juridiques permettant la rémunération des personnes qui en sont membres. En y ajoutant la garantie d'une égalité de rémunération, il vise à introduire un dispositif contraignant, alors que l'objectif du texte est de lever les obstacles au développement de l'exercice coordonné. En outre, les modalités de versement des rémunérations et de l'intéressement sont déterminées au niveau conventionnel. Il n'y a donc pas lieu d'apporter cette précision dans la loi. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable. S'agissant de l'amendement n° 787 du Gouvernement, la commission a supprimé de l'habilitation l'objectif de prévoir les conditions d'emploi et de rémunération par les maisons de santé de professionnels participant à leur mission, ainsi que des personnels intervenant auprès des médecins pour les assister dans leur pratique quotidienne. Il semble, en effet, prématuré de renvoyer à une ordonnance la question de la rémunération des assistants médicaux, alors que leur fonction, qui fait actuellement l'objet de négociations conventionnelles, n'est encore définie par aucun texte. La commission entend l'objectif du Gouvernement de n'exclure aucune des modalités d'emploi

vote sur l'amendement n° 332. L'article 19 est un article complexe, qui habilite le Gouvernement, d'une part, à simplifier les missions, l'organisation et le fonctionnement des ARS,

un amendement avait été adopté visant à autoriser à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, à déroger à l'article L. 6323-1-5 du code de la santé publique, aux termes duquel « les professionnels qui exercent au sein des centres de santé sont salariés. Cette expérimentation entre en contradiction avec un des principes fondant les centres de santé : le salariat, qui participe de l'efficacité et de la pertinence de ce mode d'exercice regroupé et coordonné.

Mme Victoire Jasmin. Cet amendement vise à étendre les pouvoirs des ARS locales, afin, notamment, de tenir compte des problématiques soulevées par les évacuations sanitaires, surtout lors de la prise en charge, tant médicale que sociale, de situations graves, comme les cancers pédiatriques. Il vise à permettre de conclure, au niveau local, des programmes de coopération sanitaire, mais aussi médico-sociale, pilotés par les ARS locales. Cette coopération décentralisée permettrait de faciliter l'accès aux soins pour les populations et de mieux coordonner l'offre de soins ou la recherche avec d'autres régions françaises

du code de santé publique, qui prévoit que « dans les territoires frontaliers et les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le projet régional de santé organise, lorsqu'un accord-cadre international le permet, la coopération sanitaire et médico-sociale avec les autorités du pays voisin.

Cet amendement tend à demander la remise d'un rapport du Gouvernement sur le financement de l'agence régionale de santé de Mayotte, qui va être créée. J'en profite pour féliciter le Gouvernement de cette mesure de justice sanitaire et sociale et pour souligner les efforts

Cette ARS profitera aux Mahorais et contribuera à lutter contre le sentiment de délaissement qui a pu s'exprimer à Mayotte ces dernières années. Sa création donnera lieu à un certain nombre de transferts et d'arbitrages financiers, pour scinder

Pour ces raisons, je souhaite faciliter la mission de contrôle du Parlement sur ce dossier, par l'intermédiaire d'un rapport dédié. Je connais la jurisprudence de notre

qui modifie les règles de composition et de vote au sein du conseil de surveillance des ARS. Plus précisément, cet article conduit à confier la présidence du conseil de surveillance des ARS à un élu

cette proposition vise à politiser la gouvernance des ARS. Je ne suis pas sûre que, dans la période actuelle, nous soyons très favorables à ce que l'État perde la main et sa capacité à veiller à l'équité entre les territoires

que certaines émanations du Gouvernement. Je rappelle d'ailleurs que le directeur de l'ARS est nommé par le Gouvernement, et le conseil de surveillance présidé par le préfet de région.

Bien qu'imparfaite, cette disposition a au moins le mérite de remettre de la représentation nationale au niveau des ARS. Elle participe du lien que nous entretenons entre nos territoires et le travail parlementaire.

médecine. Vous le savez, des négociations conventionnelles ont été ouvertes pour déterminer les conditions d'exercice et de rémunération des assistants médicaux. J'ai souhaité que ces futurs assistants médicaux aient à la fois une fonction administrative,

Mme la ministre. Cet amendement a pour objet d'harmoniser l'intitulé des plans détaillant les mesures à mettre en oeuvre en cas d'événement entraînant une perturbation de l'organisation des soins, notamment en cas de circonstances exceptionnelles,

en cas de situation sanitaire exceptionnelle, seront précisées et déclinées par voie réglementaire et d'instruction.

et mis en place à la suite des attentats de novembre 2015, semble malheureusement avoir été dévoyée ces derniers mois. Selon la CNIL, cette base de données vise à établir « une liste unique des victimes d'attentats pour l'information de leurs proches par la cellule interministérielle d'aide aux victimes » et peut être étendue à des « situations sanitaires exceptionnelles ». Or, dans le contexte du mouvement social dit des gilets jaunes, ce dispositif semble avoir été détourné par l'administration hospitalière et les agences régionales de santé, notamment l'AP-HP et l'ARS d'Île-de-France. Les autorités sanitaires ont enjoint médecins et équipes soignantes d'intégrer dans cette base de données les jaunes hospitalisés et de saisir leur identité et leurs données médicales, mais aussi tout élément d'identification physique, pour remonter des informations aux différentes autorités.

Ma chère collègue, les données inscrites dans le système d'information unique des victimes ont vocation à permettre l'identification et le suivi des victimes d'un événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle, notamment pour améliorer la prise en charge de leurs frais de santé et la coordination de leur parcours entre établissements.

745. La parole est à M. Yves Daudigny, sur l'article. Les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un État non membre de l'Union européenne contribuent au fonctionnement quotidien de nombre de services hospitaliers, en particulier dans les zones sous-dotées. Il s'agit principalement de médecins, mais aussi de chirurgiens-dentistes, de sages-femmes et de pharmaciens. Les Padhue, comme il est d'usage de les nommer, bien moins rémunérés que les autres praticiens hospitaliers et cantonnés à des contrats courts sans perspectives d'évolution, constituent pourtant une aide précieuse, quelquefois indispensable, pour nos hôpitaux.

hors de l'Union européenne. Si le règlement du sort des Padhue n'est pas aisé, c'est parce que ce statut recouvre une multitude de situations particulières. Sécuriser l'exercice de ces professionnels de santé qui interviennent chaque jour auprès de nos concitoyens est une impérieuse nécessité. L'autorisation d'exercice dérogatoire mise en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 et renouvelée trois fois, la dernière fois en décembre dernier, n'est plus tenable. L'article 21 rénove les modalités de recrutement des Padhue. Il s'agit notamment de proposer aux praticiens qui exerçaient au sein des établissements français au 31 octobre dernier de bénéficier d'une autorisation de plein exercice, sous condition d'un parcours de consolidation de compétences, afin de répondre aux exigences de la profession. L'article améliore les conditions d'intégration des Padhue dans le système de santé français et sécurise le processus de vérification des compétences acquises par la réalisation du parcours de consolidation des compétences.

au profit d'une procédure d'affectation et faire entrer les Padhue dans un processus national d'évaluation des compétences. Deux questions subsistent néanmoins. Tout d'abord, le périmètre du dispositif d'intégration doit être suffisamment large pour couvrir l'ensemble des Padhue aujourd'hui en activité ou en recherche d'activité. Ensuite, vient la question, épineuse, des binationaux titulaires d'un diplôme étranger. Ils sont très peu nombreux, mais se retrouvent dans une impasse, car ils ne satisfont

Je note dans cet amendement une discordance importante entre l'objet de l'amendement et le dispositif. Celui-ci modifie un régime d'autorisation d'exercice ancien, qui n'a plus cours

il n'existe, dans le dispositif proposé, aucune disposition établissant une quelconque différence entre les Padhue à raison de leur nationalité. Seul le lieu d'obtention

J'ai essayé de clarifier ce problème : je pense que leur demande provient très probablement d'une confusion entre plusieurs éléments. Il s'agit, semble-t-il, de praticiens qui ne satisfont pas aux conditions de la procédure d'autorisation d'exercice : cela résulte cependant non pas des textes qui leur seraient applicables à raison de leur nationalité française, mais du fait qu'ils n'ont pas suffisamment exercé au cours des dernières années. Cette absence d'exercice découle elle-même de la politique de recrutement des hôpitaux, qui se trouvent dans une zone grise dès lors que nous parlons de Padhue. Il nous est donc difficile de porter une appréciation sur ce point. Je puis en tout cas vous affirmer- Mme la ministre pourra éventuellement nous le confirmer -qu'aucune disposition inscrite à l'article 21 ne réserve l'application de la procédure d'autorisation d'exercice aux médecins de nationalité étrangère. C'est bien l'origine du diplôme qui est prise en compte.

à l'origine et la nationalité des médecins ; la seule distinction opérée l'est entre le diplôme de l'Union européenne et le diplôme hors Union européenne, quelle que soit la nationalité

amendement, dont l'initiative revient au docteur Chasseing, vise à rendre éligible à la procédure de demande d'autorisation d'exercice l'ensemble des médecins à diplôme hors Union européenne. Seuls les médecins remplissant les clauses prévues à l'alinéa 8, concernant les conditions d'activité et de durée, pourront bénéficier d'une attestation autorisant la poursuite de leur activité, dans l'attente de l'instruction de leur demande par la commission compétente,

par l'article 21, déjà élargie par la commission aux professionnels exerçant dans les établissements de santé privés et dans le médico-social, a atteint un point d'équilibre satisfaisant. Afin de garantir la qualité et la sécurité des soins dispensés aux patients, la condition d'exercice minimal et récent me paraît devoir constituer un filtre pour l'accès à la procédure d'autorisation d'exercice. trop l'accès à cette procédure, nous risquons de ralentir sa mise en oeuvre et de laisser, pendant ce temps, se reconstituer un ensemble de Padhue exerçant dans l'illégalité. L'amendement n° 635

eux seraient ainsi privés du droit de présenter leur dossier à la commission et de faire valoir leurs compétences simplement parce qu'ils n'étaient pas en poste le 31 octobre 2018.

La condition d'une présence effective entre le 1 octobre 2018 et le 31 janvier 2019 sur le lieu d'exercice conduit à exclure du dispositif des professionnels pourtant en activité dans notre système de santé depuis 2015, et pour plusieurs années, du fait, par exemple, d'une période de latence entre deux contrats, d'une formation médicale ou une reconversion professionnelle provisoire dans le domaine de la santé.

tend quant à lui à élargir la notion des dates, afin d'inclure les professionnels de santé ayant cumulé deux ans d'activité dans le système de santé depuis 2015 jusqu'en octobre 2020, date de dépôt

Nous avons en France, très certainement- sûrement, même -, des praticiens compétents et motivés qui ne peuvent exercer du fait du lieu d'obtention de leur diplôme. Si les Padhue voient leurs conditions s'améliorer grâce à l'article 21, certaines catégories de ces praticiens restent exclues du dispositif. Compte tenu des difficultés que rencontrent ces médecins pour trouver un poste, cet amendement vise à supprimer la période d'obligation de présence en établissement. Une obligation d'exercice de deux ans entre 2015 et 2017 nous semble suffisante, d'une part, au regard des restrictions très fortes qui existent actuellement et qui empêchent les Padhue de trouver un poste- certains d'entre eux ont d'ailleurs renoncé à chercher un emploi pour se consacrer pleinement à la préparation du concours -, et, d'autre part,

conditionnée à un dossier de demande validé par un comité, qui peut, par ailleurs, exiger du praticien, une remise à niveau de ses compétences.

entre 2015 et 2018, et une condition de présence, entre le 1 octobre 2018 et le 1 janvier 2019. Cette seconde condition se justifie par la préoccupation d'ouvrir la procédure d'autorisation d'exercice uniquement aux Padhue qui exercent actuellement et effectivement dans notre système de santé. Il ne faudrait pas créer un effet d'aubaine en ouvrant cette possibilité à des personnes qui auraient quitté notre territoire depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Afin d'éviter de rendre inéligibles des Padhue qui auraient connu une rupture de contrat, la commission des affaires sociales a déjà élargi cette condition de présence, en substituant un intervalle de temps à une condition de présence un jour donné. Je le rappelle, le texte qui nous a été transmis par l'Assemblée nationale prévoyait une condition de présence au 31 octobre 2018.

498 rectifié est retiré.

Si,, les Padhue actuellement en exercice devraient plutôt être en poste dans les établissements publics, sous des statuts tels que celui de médecin faisant fonction d'interne ou de praticien assistant associé, il semble que certains d'entre eux aient pu être recrutés par des établissements de santé privés. Ces situations ont été favorisées par les recrutements illicites des établissements de santé, dans un cadre général de tolérance des situations souvent inadmissibles dans lesquelles se sont retrouvés les Padhue. Il me semble pourtant que nous devons nous montrer équitables et en tenir compte.

l'exercice en clinique privée n'altère pas vos compétences en tant que médecin. Les établissements privés à but lucratif offrent les mêmes services et soins au grand public et garantissent une prise en charge complète dans un environnement plus pluridisciplinaire.

Au-delà de l'aspect juridique du statut de l'établissement, les institutions de soins à but lucratif offrent les mêmes services et les mêmes soins au grand public et garantissent la même prise en charge médicale dans un univers pluridisciplinaire.

l'amendement n° 781 rectifié, il est nécessaire que les conseils départementaux de l'ordre des médecins connaissent les médecins concernés par cette nouvelle procédure et qui exercent sur leur territoire, afin de satisfaire à l'obligation d'information auprès des médecins et des patients.

la commission nationale d'autorisation d'exercice ne saurait émettre un avis sans avoir auparavant auditionné le candidat. En outre, dans l'hypothèse d'un défaut de compétence, il est essentiel que cette commission auditionne le candidat afin de définir le parcours de consolidation. Quel est l'avis de la commission ? La

mais une seule commission d'autorisation d'exercice à l'échelle nationale. Celle-ci existe déjà aux termes de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. La composition de cette commission nationale est précisée

paraît satisfaisant à la commission : seuls seront auditionnés au niveau national les candidats qui pourront directement accéder au plein exercice et ceux qui verront leur demande rejetée. La commission aura cependant la possibilité d'auditionner les autres candidats dont le profil nécessiterait une investigation approfondie. Ces autres candidats auront, par ailleurs, vu leur dossier préalablement examiné par la commission régionale. une audition obligatoire de tous les candidats conduirait au ralentissement de la procédure et viderait probablement de son sens la pré-instruction des dossiers au niveau régional. En conséquence, nous demandons le retrait de

en établissement de santé, et permettra de régulariser un grand nombre d'entre eux. Pour autant, elle ne permet pas de régler la situation de l'ensemble des Padhue. Il n'est bien entendu pas souhaitable d'ouvrir trop largement la procédure temporaire prévue par l'article 21, et ce pour deux raisons

Certaines situations paraissent cependant devoir être prises en compte. C'est par exemple le cas des Padhue qui ont exercé, non pas directement auprès des patients, mais dans une agence de santé telle que la Haute Autorité de santé, la HAS, où ils ont rendu de grands services à notre système de santé. Je pense également à ceux qui ont interrompu leur activité professionnelle pour préparer le concours exigeant de la liste A et s'inscrire ainsi dans la légalité. Pour ces profils particuliers, je propose non pas d'élargir les conditions de la procédure d'autorisation d'exercice dérogatoire, mais de faire préexaminer leur dossier par la commission nationale d'autorisation d'exercice, qui leur permettra ou non de se rattacher à la procédure d'autorisation d'exercice dérogatoire. Il s'agit donc uniquement de leur donner ou non accès à cette procédure.

n'est véritablement satisfaisante au vu de la diversité des profils des Padhue et des situations d'illégalité dans lesquelles ils sont cantonnés, cette mesure permettrait au moins de répondre à certaines situations particulièrement injustes.

Comme je l'ai déjà souligné à plusieurs reprises, il est indispensable de fixer des conditions objectives permettant de préserver la qualité des soins et de réserver la procédure aux Padhue effectivement intégrés dans notre système de santé. Cela aboutit nécessairement à exclure certains praticiens du fait, le plus souvent, de parcours de vie accidentés. C'est regrettable, mais inévitable. Je dois cependant dire que j'ai été sensible à la situation individuelle de certains de ces praticiens. Je pense notamment à toutes ces personnes qui exercent actuellement au sein d'agences de santé,

à certains Padhue dont la spécialité ne figure pas au concours de la liste A et qui, pour des raisons diverses, n'ont pu se rattacher à la condition d'exercice. Faute de recensement des Padhue actuellement présents sur notre territoire et dans notre système de santé, il est difficile d'évaluer si ces situations sont nombreuses ou résiduelles. De ce fait, je ne souhaite pas trop élargir la procédure d'autorisation d'exercice prévue par l'article 21.

Comme notre collègue Fabien Gay l'a souligné, nous avons eu l'occasion de rencontrer des professionnels de santé diplômés d'États non membres de l'Union européenne, naturalisés Français, qui ne peuvent exercer leur art, faute de places ouvertes au concours. Actuellement, pour exercer en France, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires d'un diplôme obtenu dans un pays non membre de l'Union européenne doivent, en principe, principe, obtenir une autorisation de plein exercice grâce à la procédure de droit commun dite de la liste A. Selon cette procédure, les praticiens doivent réussir un concours comportant des épreuves de vérification des connaissances et justifier d'un niveau de maîtrise suffisante de la langue française. Les praticiens ayant la qualité de réfugié, d'apatride, de bénéficiaire de l'asile territorial ou de la protection subsidiaire, ainsi que les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités des autorités françaises en considération de la situation de crise dans leur pays de résidence bénéficient d'une procédure dérogatoire d'autorisation sur examen, dite de la liste B : le nombre maximal de candidats susceptibles d'être reçus au concours de la liste A ne leur est pas applicable. Enfin, le dispositif dérogatoire dit de la liste C accorde à certains praticiens une autorisation temporaire d'exercer et la possibilité de passer un examen spécifique pour l'obtention d'une autorisation de plein exercice. Notre amendement vise à autoriser les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen de passer le concours de la liste A. proposé par Mme Gréaume me paraît discriminatoire vis-à-vis des Padhue extra-européens Par ailleurs, je pense qu'il n'est pas souhaitable de laisser des personnes dans l'expectative pendant de très nombreuses années. Je souligne enfin que le nombre de places au concours dit de la liste A

souhaitons que le patient puisse donner à l'établissement de santé au sein duquel il est hospitalisé les coordonnées du professionnel de santé de son choix, afin d'organiser la continuité des soins et sa sortie, comme le prévoit l'article L. 1111-2 du code de la santé publique.

permettent d'accompagner des personnes en situation de précarité, sans hébergement stable, et atteintes d'une pathologie chronique. L'intervention des équipes d'accompagnement des ACT sous la forme de services fait depuis plusieurs années l'objet d'expériences locales et d'une expérimentation nationale pour cinquante places. Cet amendement vise à étendre ce dispositif à l'ensemble des départements. Les interventions dans les

un peu moins de passion ! Depuis une ordonnance du 26 janvier 2005, un dispositif spécifique permet au directeur général de l'agence régionale de santé de Guyane

rapport établi toujours en 2017 par le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, dénonce également les déserts médicaux à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon. La situation est encore plus préoccupante si l'on considère l'âge des médecins en exercice aujourd'hui. En effet, le syndicat des médecins généralistes de France souligne que, compte tenu des départs à la retraite, la moitié des cabinets de médecins généralistes devrait fermer dans les cinq prochaines années

avant que le nouveau président brésilien Jair Bolsonaro y mette fin au début de cette année, obligeant les 8 000 médecins cubains exerçant au Brésil à quitter le pays. Pourtant, nous savons tous que ces médecins sont reconnus internationalement. Je tiens à souligner l'importance de cette mesure tout en rappelant que les conditions requises, très strictes, peuvent rendre difficile le recrutement effectif des médecins. En Guyane, alors que cette mesure a été adoptée en 2005, elle reste peu appliquée, l'ordre des médecins de Guyane y étant généralement hostile.

territoires d'outre-mer et, singulièrement à la Guadeloupe et à la Martinique, des autorisations temporaires d'exercice pour les praticiens diplômés dans un État non membre de l'Union européenne.

en Guyane, le représentant de l'État peut autoriser, par arrêté, un médecin titulaire d'un diplôme de médecine, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans la région.

confrontés à une désertification médicale de plus en plus problématique : difficultés de recrutement, pression démographique, manque d'attractivité. Avec le présent amendement, nous allons plus loin tout en visant les mêmes objectifs : sécuriser et élargir. d'étendre le dispositif à d'autres professions : chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien. Par ailleurs, une commission territoriale d'autorisation d'exercice devra émettre un avis préalablement à la délivrance de toute autorisation d'exercice par arrêté du directeur général de l'ARS concernée. Cette autorisation d'exercice est temporaire et circonscrite à l'exercice au sein du territoire visé et dans les structures de santé. Le nombre de professionnels autorisés

Quel est l'avis de la commission ? La commission s'est prononcée en faveur de l'extension à la Martinique et à la Guadeloupe du dispositif dérogatoire d'accès à l'autorisation d'exercice en vigueur en Guyane, afin de répondre à l'insuffisante densité du maillage sanitaire sur ces territoires. Ce dispositif permet au directeur général de l'ARS d'autoriser, par arrêté, un médecin étranger ou titulaire d'un diplôme de médecine obtenu hors Union européenne à exercer dans la région. vise à préciser la procédure applicable à ce dispositif dans le cadre de son extension aux Antilles.

d'harmoniser et d'améliorer le dispositif dans les collectivités concernées par la dérogation, y compris à Saint-Pierre-et Miquelon où le préfet est compétent pour accorder cette dérogation. Il vise par ailleurs à étendre le dispositif aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes, ainsi qu'aux pharmaciens. Il limite le champ de la dérogation aux structures de santé et la limite également dans le temps, puisqu'il prévoit une application jusqu'au 31 décembre 2025. Il a pour objet d'établir enfin deux commissions territoriales d'autorisation d'exercice, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, afin de garantir un recrutement de qualité,

La commission n'a pas pu examiner le sous-amendement n° 833 rectifié, compte tenu de son dépôt tardif. C'est donc à titre personnel que j'émettrai un avis. Il me semble que ce sous-amendement est satisfait par l'amendement n° 604, puisque Saint-Martin est dans le ressort de l'ARS de la Guadeloupe. Je m'en remettrai toutefois à l'avis du Gouvernement

Mme la ministre. Le présent amendement vise à répondre à une mise en demeure de la Commission européenne sur la transposition de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Il s'inscrit dans le cadre des échanges qui ont eu lieu entre les autorités françaises et la Commission européenne.

a pour objet de répondre à un grief de la Commission européenne qui considère que les modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles des opticiens-lunetiers en France ne seraient pas conformes aux exigences de la directive.

Mme la ministre. Cet amendement vise à adapter aux collectivités de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie certaines dispositions, notamment l'hébergement de données à caractère personnel et les modalités d'organisation de soins psychiatriques.

L'amendement n° 44 rectifié tend à rééquilibrer la réforme de la procédure d'évaluation sociale et médico-sociale introduite par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Il s'agit de permettre à une association gestionnaire de rédiger des observations

En effet, le fait de définir et de qualifier ce qui est de la communication à caractère promotionnel relative aux plasmas et, donc, par définition, ce qui n'entre pas dans ce champ permet de positionner l'Établissement français du sang- ou EFS -par rapport à des concurrents privés. Je pense particulièrement à Octapharma.

souci d'alerter sur le risque de voir des produits dérivés du sang, issus de laboratoires privés, pénétrer au sein des hôpitaux publics, sans qu'il n'y ait aucun dispositif de traçabilité de l'origine des poches de plasma. On le sait, le service public du sang, dont l'EFS est le garant, est mis à mal depuis plusieurs années par des intérêts financiers qui voient la commercialisation des produits sanguins comme une affaire extrêmement rentable, là où les questions d'éthique, de traçabilité et de sécurité sanitaire devraient l'emporter. Je profite de cette intervention pour vous demander, madame la ministre, un point sur la situation du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies- le LFB -, qui était jusqu'ici détenu à 100 % par l'État français et dont le capital vient d'être ouvert. Comment comptez-vous continuer à assurer que les principes fondateurs de la filière sang et l'accès des patients aux médicaments dérivés du sang ne soient aucunement affectés par cette évolution ? Je vous remercie, par avance, de votre réponse.

Cet amendement vise à permettre aux usagers de participer aux instances disciplinaires des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes. Il s'agit d'une demande récurrente des associations d'usagers, laquelle, nous semble-t-il, peut s'entendre. Nous avons donc souhaité

particulièrement en cas d'abus sexuel, lequel est d'ailleurs considéré comme une circonstance aggravante par les juridictions. Des modes d'information entre les juridictions disciplinaires et le procureur de la République sont déjà prévus. Aussi, si le sujet est grave et mérite d'être traité avec toute l'attention nécessaire, cet amendement paraît satisfait.

: La parole est à M. Dominique Théophile. Cet amendement tend à réviser la composition du Conseil national de l'ordre des médecins, tel qu'il sera renouvelé en 2022. Il s'agit de prévoir trois binômes pour représenter l'interrégion Antilles-Guyane au Conseil national de l'ordre pour ajuster sa représentativité,

entre régions ultramarines. La représentation du conseil interrégional Antilles-Guyane passerait de deux à trois binômes, soit le même niveau que celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes, alors que les populations des régions concernées s'inscrivent dans un rapport de un à La Réunion et Mayotte demeureraient représentées, quant à elles, par un seul binôme. Nous pouvons toutefois comprendre la volonté de renforcer la représentation de l'interrégion Antilles-Guyane, au regard notamment des règles qui prévalaient avant l'ordonnance du 16 février 2017

d'accroître la représentation des médecins d'outre-mer dans le Conseil national de l'ordre. Une telle disposition aurait pour conséquence de faire passer de 56 à 58 le nombre de membres siégeant au Conseil national, mais elle entraînerait certainement une surreprésentation des outre-mer,

Imbert, pour présenter l'amendement n° 6 rectifié . Le code de la santé publique prévoit que « les pharmaciens exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement, ou aux rapports entre associés La problématique ordinale, indépendamment du financement envisagé, est de vérifier que le financement dont pourrait bénéficier le pharmacien n'entrave pas son indépendance professionnelle. Afin que l'Ordre des pharmaciens puisse apprécier, justement, le respect de cette condition, il est nécessaire que lui soient communiqués également les conventions et avenants relatifs rapports entre associés et intervenants concourant au financement de l'officine ou du laboratoire de biologie médicale. La parole est à Mme Viviane Malet,

La prise d'un décret suffirait. Ce décret pourrait en outre avoir un caractère transversal aux sept ordres professionnels, ensuite libres d'y recourir ou non.

Aujourd'hui, le délai légal est fixé à deux ans. Le directeur général de l'ARS, dûment informé d'une reprise en cours d'une officine pourrait accorder un délai complémentaire de remplacement dans le cadre de la gérance après décès, lequel pourrait être fixé à un an maximum, afin de garantir la réalisation de la reprise. À défaut pour le repreneur de n'avoir pu faire enregistrer sa déclaration d'exploitation au terme du délai de deux ans, ou de trois ans en cas de prolongation, l'officine devra être fermée pendant un an à l'issue du remplacement sans que cette caducité ne soit constatée d'office. En définitive, l'adoption de cet amendement permettrait d'augmenter la durée maximale d'existence de la licence de trois à quatre ans après le décès du titulaire d'officine, dans le cas d'une procédure de vente en cours.

Gouvernement ? Ces amendements sont déjà satisfaits par les dispositions actuelles de la réglementation qui visent à tenir compte de ces situations particulières. Ainsi, le délai de gérance d'une officine par un pharmacien autorisé par le directeur général de l'ARS après le décès du titulaire peut aujourd'hui être de deux ans. Il fait suite pendant lequel la gérance peut être accordée à un pharmacien remplaçant lorsque l'absence du pharmacien titulaire se justifie par son état de santé. Enfin, je rappelle que les héritiers peuvent conserver l'officine pendant un an avant que la cessation définitive d'activité ne soit constatée par l'ARS.

à des cadeaux, de sorte que cette liste soit le moins possible sujette à interprétation. Les avantages commerciaux sont autorisés, pour les médicaments remboursables, sous réserve qu'ils respectent les plafonds de remises imposés par le code de la sécurité sociale.

786 rectifié , qui met l'accent sur une différence de traitement entre les étudiants en formation et les professionnels en exercice. Elle souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur cette disposition, qui relève, à l'origine, de son initiative et a été modifiée en commission par un amendement du groupe La République En Marche.

plan de contrôle de la formation continue des professionnels de santé. De plus, cette agence sera habilitée à contrôler la capacité des organismes à dispenser des formations professionnelles continues. Un décret organisera les modalités de sanction en cas de

corriger une incohérence quant à la durée des mandats des assesseurs des sections des assurances sociales des ordres des masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers et pédicures-podologues. Ces derniers sont nommés pour six ans. Or les autres membres de ces conseils sont, eux, renouvelables par moitié tous les trois ans. Aussi, un assesseur qui ne serait plus membre du conseil pourrait conserver son mandat d'assesseur à la section des assurances sociales.

pour explication de vote.

Il s'agit ainsi de renforcer la transparence du secteur et des liens que les laboratoires pharmaceutiques entretiennent avec les organismes chargés de la formation continue des professionnels de santé.

Elle doit désormais jouer pleinement son rôle dans la formation des futurs médecins de la région. Actuellement, nos étudiants partent vers l'Hexagone à partir de la quatrième année, afin de poursuivre leur parcours.

et le moment est opportun pour la mener. Toutefois, le Gouvernement ayant déjà engagé des travaux en ce sens, il n'est pas utile d'inscrire une demande de rapport dans la loi. C'est pourquoi la commission des affaires sociales a supprimé l'article 26. Elle est par conséquent défavorable à son rétablissement.

les étudiants en médecine issus des outre-mer sont accueillis par des universités de l'Hexagone, qui éprouvent déjà bien des difficultés à intégrer ce surnombre d'étudiants du fait même de l'accroissement de leur propre. Ainsi, Ainsi, en raison de la rupture entre les premier et troisième cycles et en l'absence d'accompagnement pédagogique et financier suffisant, les jeunes médecins issus des outre-mer ont tendance à ne pas y revenir pour s'y installer, faute de perspectives de spécialisation ou de carrière hospitalo-universitaire attractive. Il s'agit, par cet amendement, de maintenir le lien avec l'université d'origine en donnant à cette dernière les moyens de rattrapage vis-à-vis des autres universités de l'Hexagone, notamment en développant l'usage des nouvelles technologies et la coopération sur des sujets de recherche spécifiques à ces régions. Quel

nous demandons la remise d'un rapport sur les perspectives de transformation du groupement hospitalier de territoire de Guyane en un centre hospitalier universitaire. a été pris acte de la création du groupement hospitalier de territoire de Guyane, le GHTG. Celui-ci regroupe le centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne, celui de Kourou, ainsi que celui de l'ouest guyanais Franck Joly. Ensemble, les trois établissements publics de santé de Guyane seront plus forts pour développer leur offre de soins et être plus attractifs. Nous le savons, monsieur le rapporteur, vous allez émettre un avis défavorable sur cette demande de rapport, conformément à la position traditionnelle de la commission sur ce type d'amendement. plus ne sommes pas friands de rapports. Toutefois, nous pensons qu'il est important d'avoir ce débat aujourd'hui et de réfléchir à cette question pour trouver à terme des solutions pérennes et efficaces, afin de désengorger le système de santé de la Guyane et de renforcer son attractivité. Depuis le début de l'examen de ce texte, nous parlons de déserts médicaux. De par leur situation démographique, leur enclavement et leur géographie, la Guyane et les outre-mer en général- nous avons évoqué longuement le cas de Mayotte -sont extrêmement -sont extrêmement touchés par la désertification médicale. Dans ce contexte, le GHTG qui vient d'être créé a vocation à devenir un CHU à part entière. Cette transformation a plusieurs objectifs : meilleur recrutement de personnel, développement des unités de recherche sur les pathologies infectieuses et tropicales,

de saluer la présence, dans notre tribune officielle, d'une délégation de sénateurs et de sénatrices, membres du Congrès américain, conduite par M. Johnny Isakson, président de la commission sénatoriale de la déontologie ainsi que de celle des anciens combattants. La délégation effectue actuellement un séjour en France à l'occasion du soixante-quinzième anniversaire du débarquement de Normandie. Elle a été reçue ce matin par notre collègue, M. Christian Cambon, président M. Christian Cambon, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, accompagné de membres de la commission, ainsi que par M. Antoine Lefèvre, président du groupe interparlementaire d'amitié France-États-Unis et certains membres du groupe. Cette rencontre a donné lieu à un échange fructueux sur l'état de la relation transatlantique, notamment en matière de sécurité, en Europe et au Moyen-Orient, ainsi que dans les domaines économiques et commerciaux. Nous sommes particulièrement sensibles à cette visite qui nous permet de renouveler, à l'occasion des commémorations du débarquement, la profonde amitié qui lie nos deux pays, dans le cadre des relations anciennes anciennes et fructueuses entre nos deux assemblées, si bien rappelées hier par le président Gérard Larcher. Au nom du Sénat de la République, je souhaite à la délégation la plus cordiale bienvenue et je forme des voeux pour que son séjour en France soit profitable et contribue à approfondir les liens qui unissent nos deux pays. Nous

Nous voulons en effet savoir ce qu'il en est exactement de l'usage par les médecins de la clause de conscience spécifique et des inégalités territoriales.

au combat entre les anti-IVG et les pro-IVG, puisque, depuis le début, les anti-IVG n'ont cessé de multiplier les obstacles. Les inquiétudes sont aussi renforcées par la

ou le désintérêt d'un certain nombre de praticiens, de jeunes internes, de jeunes médecins, qui pensent qu'il ne s'agit pas d'un acte médical noble grâce auquel ils vont pouvoir mener une belle carrière hospitalière. C'est pourquoi je m'apprête

or on ne peut pas se reposer sur les autres ni être à la merci des législations de ces pays. Après discussion avec de nombreux professionnels de santé,

Le véritable enjeu, me semble-t-il, réside donc moins dans le réexamen de ce délai que dans les efforts qui doivent être faits pour prévenir les situations d'urgence. À cet égard, la bonne information des patientes est fondamentale. Une fois leur décision prise, il est capital qu'elles puissent engager les démarches rapidement, car les délais de prise en charge peuvent en effet être longs dans certaines régions. Des progrès ont été réalisés pour réduire ces délais en facilitant l'orientation des patientes vers des structures pertinentes sur le territoire. Depuis l'adoption de la loi Touraine, certains centres de santé peuvent ainsi

de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la Drees. Depuis l'adoption de la loi du 17 janvier 1975, dite loi Veil, l'accès à l'IVG reste difficile, voire l'est de plus en plus.

ailleurs, l'article L 2212-8 du code de la santé publique prévoit que, au-delà de la clause de conscience générale s'appliquant aux médecins pour tout acte médical, l'IVG est concernée par une clause de conscience spécifique. Des exemples récents, notamment l'absence d'IVG à l'hôpital du Bailleul à La Flèche, faute de médecins, et les propos tenus par le président du Syndicat national des gynécologues et obstétriciens ont montré que le recours à cette double clause est important et peut, dans un contexte de pénurie de médecins et de structures, constituer un obstacle supplémentaire. Qui plus est, cette

En France, la clause de conscience spécifique, je le rappelle à tous mes collègues, s'ajoute à la clause de conscience générale prévue dans le code de déontologie, qui garantit à tous les soignants la possibilité de refuser de faire un acte médical avec lequel ils seraient en désaccord. Cette clause de conscience spécifique, qui n'existe que pour l'IVG, stigmatise cet

vous avez fait campagne voilà quelques semaines en reprenant la clause de l'Européenne la plus favorisée, qui avait été élaborée par Gisèle Halimi. Vous avez proposé un bouquet législatif pour les femmes en Europe,

puisqu'un médecin pourrait toujours refuser, en application de la clause de conscience générale, de pratiquer une IVG, mais n'aurait plus, dans la configuration proposée par le biais des amendements n 349 et 735 rectifié l'obligation de rediriger la patiente vers un autre professionnel ou une autre structure. de l'amendement n° 735 rectifié ne parvient pas à préserver cette obligation pour tous les praticiens, dans la mesure où il tend à insérer une précision sur l'obligation de réorientation au troisième alinéa de l'article L. 2212-18 du code de la santé publique, ce qui n'est pas suffisant, car cet alinéa ne vise que les IVG pratiquées en établissement privé, alors même que les femmes en situation de détresse sont majoritairement prises en charge dans le secteur public. Enfin, l'amendement n° 630 rectifié est problématique sur le plan constitutionnel. En effet, la mise en place de sanctions pour ce qui concerne la carrière, notamment par des licenciements ou rétrogradations, en cas d'exercice de la clause de conscience générale ne semble pas compatible avec la liberté de conscience garantie à tout citoyen par la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme.

Je comprends votre argumentaire, madame Rossignol, il est limpide et coule de source. Il faut par principe ne pas stigmatiser le droit

Le scrutin est ouvert.

des responsabilités d'un médecin obstétricien, de l'approche globale de la santé reproductive des femmes. On ne peut pas être pour la

de faire en sorte que cet acte d'interruption volontaire de grossesse fasse partie du droit commun.